Il avait initialement pour objet de supprimer l'avis consultatif de la commission administrative paritaire en matière d'avancement et de promotion interne dans chaque versant de la fonction publique. Il était de rendre obligatoire l'élaboration de lignes directrices de gestion pour déterminer la stratégie annuelle de pilotage des ressources humaines, des lignes qui seront désormais opposables à l'administration et sur lesquelles les nouveaux comités sociaux seront consultés. Nous sommes favorables à l'élaboration de telles lignes de gestion, qui vont amener un cadre bienvenu, ainsi que de la transparence. Nous sommes, à l'inverse, vous l'aurez compris, absolument défavorables à la dévitalisation des instances de dialogue social qui mettent quotidiennement en oeuvre le principe de participation des fonctionnaires. Ce principe veut que les agents soient associés aux mesures qui les concernent, que celles-ci soient individuelles ou collectives. Il est l'application à la fonction publique du principe posé par le préambule de la Constitution de 1946, en vertu duquel tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises », principe dont le Conseil constitutionnel a affirmé l'application à la fonction publique dès 1977. Cette participation des fonctionnaires est mise en oeuvre, selon l'article 9 du statut général, « par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organes consultatifs ». Nous sommes ainsi satisfaits, en vertu de ces principes, que la commission ait rétabli les CAP dans leurs rôles relatifs à la promotion et à l'avancement, tout en conservant l'apport de lignes directrices. Reste que nous sommes encore au milieu du gué, puisque cet avis demeure supprimé pour les mutations et la mobilité des fonctionnaires. Nous portons donc sur cet article 14 le même regard que sur l'article 4 de ce projet de loi, et nous voterons contre. La parole est à M. Jérôme Durain, sur l'article. Par cohérence avec les amendements de suppression que nous avions déposés sur l'article 1 et nous avons l'intention de continuer à combattre cette dévitalisation du dialogue social, puisque nous estimons que tel est aboutissent plusieurs articles de ce projet de loi, notamment dans la dimension des lignes de gestion. Ces lignes peuvent certes être un cadre général auquel l'employeur public associe les représentants des des agents publics. Toutefois, elles ne sauraient en aucun cas constituer une contrepartie à l'affaiblissement des instances de participation et de dialogue social mises en oeuvre par d'autres articles du projet de loi. Nous ne souscrivons pas à l'idée selon laquelle les agents publics ne seraient plus consultés, via les instances de dialogue social, sur les décisions personnelles relatives aux carrières. La consultation se réduirait dorénavant aux comités sociaux

Pour résumer notre sentiment, le comité social ne remplacera les CHSCT. Le seul discernement de l'employeur public ne remplacera pas le rôle de la CAP. Et les lignes directrices de gestion ne remplaceront pas le dialogue social

que l'avis de la CAP permet d'encadrer l'appréciation par l'administration de la valeur professionnelle de ses agents. La CAP est également un lieu d'échange avec les représentants du personnel, qui permet à l'employeur public de justifier la manière dont il a apprécié les dossiers et procédé au classement. Ce rôle est particulièrement important en matière de promotion interne dans les communes et établissements publics affiliés à un centre de gestion. La liste d'aptitude est, dans ce cas, établie par le président du centre de gestion, et seul le passage en CAP vient légitimer le classement opéré, tant aux yeux des collectivités qu'aux yeux des agents. La commission a maintenu les lignes directrices les lignes directrices de gestion, non plus pour se substituer à l'avis de la CAP, mais pour servir de guide lors de l'élaboration des tableaux et listes par l'employeur public, guide dont la CAP pourrait ensuite vérifier la bonne application. C'est la raison pour laquelle j'émets, au nom

Nous ne sommes pas défavorables aux lignes directrices de gestion, qui peuvent constituer une doctrine en matière de promotion ou de gestion des ressources humaines. Pour autant, cela n'exclut pas

le traitement des questions individuelles dans les CAP favoriserait le cloisonnement, le corporatisme et une gestion des ressources humaines excessivement égalitaire et uniformisatrice.

Ce sont des avis, qui garantissent, effectivement, la transparence et l'acceptabilité des décisions. Nous trouvons tout à fait dommageable que ces lignes directrices de gestion se substituent totalement aux pratiques antérieures

administration, devront prendre en compte les problématiques démographiques et les caractéristiques spécifiques des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires.

voie, aspirent désormais à servir leur collectivité d'origine. prendre en compte les problématiques démographiques et les caractéristiques spécifiques des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. sont originaires. Il s'agit de veiller à ce que les politiques mises en place dans les trois fonctions publiques prennent en considération les problématiques spécifiques à ces collectivités, en s'assurant,

Victorin Lurel, vise à ce que les lignes directrices de gestion soient déclinées au sein de chaque collectivité relevant de l'article 72-3 de la Constitution, Plus précisément, son objet est de veiller à ce que les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours intègrent les problématiques propres à chacune des collectivités d'outre-mer. amendement vise également à mettre en place un dispositif, géré par le préfet ou l'autorité déconcentrée équivalente, permettant de coordonner au niveau du territoire la mobilité et les politiques de valorisation des parcours et des compétences entre les différents services et les différentes fonctions publiques. Ce dispositif de coordination permettrait de favoriser les carrières professionnelles locales, notamment pour les cadres de la fonction publique de l'État, et d'éviter des allers-retours fréquents entre l'outre-mer et la métropole. Cet objectif de priorité donnée au recrutement local de cadres ultramarins nécessiterait le renforcement de l'interministérialisation de la gestion des effectifs outre-mer et la création d'une sorte de CAP territoriale outre-mer, ainsi que l'avait recommandé le député Patrick Lebreton

afin qu'elles fassent l'objet d'une coordination transversale aux trois fonctions publiques et incluent un dispositif de priorisation des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant le centre de leurs intérêts matériels et moraux.

Cet amendement vise en effet à rétablir les dispositions initiales du projet de loi relatives à la suppression des compétences des CAP en matière d'avancement et de promotion. Nous avons évoqué ce sujet assez longuement précédemment ; c'est l'un des points de désaccord les plus importants entre les dispositions adoptées par votre commission et les objectifs du Gouvernement.

les préoccupations de leurs auteurs semblent de nouveau porter sur les lignes directrices de gestion en matière de mobilité ; ils souhaitent notamment prendre en compte le centre des intérêts matériels et moraux dans le cadre des politiques de mobilité. Cette préoccupation semble être satisfaite au niveau réglementaire, dans le cadre du décret d'application attendu à l'article 11. Par ailleurs, je ne pense pas que les lignes directrices de gestion soient de bons outils pour mettre en place une politique à l'échelle nationale, car elles sont destinées à être conçues par chaque employeur public, au plus près de ses besoins spécifiques en matière de ressources humaines, en fonction des caractéristiques de sa structure. Je demande donc à leurs auteurs de

dans la mesure où celles-ci sont conçues comme des barèmes ou des outils d'aide à la décision. Les employeurs publics restent maîtres de leur classement, dès lors qu'ils sont capables de justifier auprès de la CAP qu'ils ont respecté les indications de ces lignes directrices.

satisfait. Quant à l'amendement n° 292 rectifié , la question des quotas fixés annuellement est complètement indépendante des lignes directrices de gestion, qui portent sur une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Les quotas sont évalués chaque année,

! Les quotas sont connus chaque année, mais les lignes directrices de gestion peuvent être déterminées pour plusieurs années. On n'est pas obligé de revenir sur les lignes directrices de gestion chaque année. Les deux sont complètement indépendants : les lignes n'ont pas à fixer les quotas.

Les lignes directrices de gestion n'ont pas de valeur légale. Elles sont arrêtées par les comités sociaux d'établissements territoriaux ou d'administrations. Elles sont invocables en cas de recours ; en cela, je partage l'avis de Mme la rapporteur sur l'amendement n° 292 rectifié . La priorité

Pour justifier ce transfert, nos rapporteurs ont indiqué que l'insuffisance professionnelle n'induisait pas de faute caractérisée de l'agent, mais « un manque de diligence, de rigueur dans l'exécution du travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles qui est préjudiciable à la bonne marche du service ». l'insuffisance professionnelle se distingue d'une faute disciplinaire et ne peut donner lieu à sanction. Reste tout de même qu'elle peut justifier un licenciement. Nous ne croyons pas que le fait que le fonctionnaire soit compliqué devant un conseil de discipline implique qu'il ait commis une faute disciplinaire. Le renvoi de ces questions au conseil de discipline tient plutôt, à nos yeux, à la formation spécifique de ce dernier et aux garanties attachées à cette procédure, qui est très particulière : l'autorité administrative doit constituer un dossier disciplinaire

L'administration doit procéder à la communication du dossier en adressant au fonctionnaire une lettre précisant qu'une procédure disciplinaire est envisagée à son encontre et présentant les griefs retenus et la sanction envisagée. La lettre doit préciser par ailleurs que l'agent peut consulter son dossier administratif, qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et qu'il peut présenter ses observations sous un délai défini.

l'amendement n° 393. Le Gouvernement a porté un regard très favorable sur bien des dispositions adoptées par votre commission des lois en matière disciplinaire ou pour les fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Nous aurons l'occasion de nous exprimer sur d'autres aspects ; je pense notamment aux questions relatives à la grève. Concernant les dispositions relatives au licenciement pour insuffisance professionnelle, nous considérons que sortir du champ du conseil de discipline cette question pour l'intégrer dans celui de la CAP est peut-être un peu rapide. C'est pourquoi nous proposons la suppression de

La commission a souhaité réintégrer le licenciement pour insuffisance professionnelle dans les compétences de la CAP en formation ordinaire, comme cela a été expliqué. Il faudrait tout Il faudrait tout de même suivre une procédure adaptée. Le fonctionnaire concerné serait convoqué à un entretien préalable avec son supérieur hiérarchique, et non plus devant un conseil de discipline. À notre sens, l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute disciplinaire, et un traitement disciplinaire nous paraît inapproprié.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

L'article 15 élargit le choix des sanctions disciplinaires et harmonise l'échelle des sanctions entre les trois versants de la fonction publique. Il supprime également les dispositions précisant la composition des CAP siégeant en conseil de discipline dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Concrètement, cette harmonisation se traduit non par un allégement des sanctions, mais par une aggravation et un alignement sur le versant de la fonction publique le plus sévère. Ainsi, dans la fonction publique territoriale est instaurée une exclusion temporaire de trois jours en sanction du premier groupe. Or, d'après la direction générale de l'administration et de la fonction publique, les sanctions les plus fréquemment prononcées par les ministères en 2017 ont justement été des sanctions de cette catégorie : elles représentent 80 % des mesures prises par les ministères à l'encontre de fonctionnaires. Nous pouvons donc légitimement craindre un recours plus important à des exclusions temporaires pour les fonctionnaires territoriaux, sanctions qui portent de lourdes conséquences pour ces agents puisque, lors d'une période d'exclusion temporaire de fonctions, le fonctionnaire est écarté du service et ne perçoit aucune rémunération. Il perd également ses droits à l'avancement d'échelon et de grade et ses droits à la retraite. Par ailleurs, les jours d'exclusion sont aussi déduits pour le calcul de ses droits au congé annuel. Ce n'est donc ni une bagatelle ni une sanction symbolique, comme le laissaient entendre les rapporteurs. La commission a même renforcé la sévérité de ces sanctions, puisqu'elle a permis la révocation dès qu'une deuxième exclusion temporaire de fonctions intervient, quel qu'en soit le groupe. Une exclusion de trois jours pourrait ainsi entraîner la révocation du sursis d'une exclusion de sept jours. Par ailleurs, la commission a obligé le conseil de discipline à motiver

madame la présidente. Quel est l'avis de la commission ? commission a en effet renforcé le régime disciplinaire applicable aux trois versants de la fonction publique en supprimant la restriction introduite par le Gouvernement en matière d'abaissement d'échelon ou de dégradation,

secrétaire d'État. Il s'agit de permettre aux personnes citées comme témoins dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estiment victimes d'actes de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes de la part de l'agent qui fait l'objet de l'action disciplinaire de demander au président de la juridiction de bénéficier de l'assistance de la tierce personne de leur choix.

les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale et modifiées par la commission des lois du Sénat, à savoir les règles relatives à l'abaissement d'échelon et à la rétrogradation, l'absence de volonté de durcissement des conditions de sursis en cas d'exclusion temporaire, la confirmation du maintien de la parité numérique dans les conseils de discipline de la fonction publique territoriale.

-de moins de trois jours. Actuellement, la révocation du sursis n'est possible qu'en cas de prononcé d'une sanction du deuxième ou troisième groupe. Avec cette disposition, la commission des lois assimile l'ETF de trois jours à une sanction du deuxième ou troisième groupe. Or la commission des lois

en permettant aux représentants du personnel d'un grade inférieur d'y siéger. Or, selon un principe général du droit, seuls les fonctionnaires ayant des grades équivalents à celui de l'agent pour lequel le conseil de discipline se réunit peuvent y siéger. Il est donc indispensable que ce principe demeure appliqué dans les conseils de discipline. Quel est l'avis de la commission

Les syndicats que nous avons rencontrés ont appelé notre attention sur les conséquences de cette exclusion temporaire dans la vie des agents en l'absence de commission de discipline, allant parfois jusqu'à décrire des situations extrêmement graves, par exemple, dans certaines professions, des suicides d'agents qui se sentent un peu abandonnés et, d'une certaine manière,

La généralisation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours au titre des sanctions du premier groupe signifie que cette sanction pourra être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. Il s'agit donc de mettre face à face un agent et son supérieur hiérarchique. Or, dans certaines

assurée que par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. Le fonctionnaire ne bénéficierait ni de la possibilité d'être entendu pour sa défense par l'organisme paritaire ni de la faculté de saisir en révision de la sanction la commission de recours. Pourtant, il s'agit d'une sanction extrêmement lourde dans la mesure où elle peut conduire à priver le fonctionnaire concerné d'une partie de sa rémunération allant jusqu'à 10 %. Cet amendement vise donc à renforcer les garanties offertes au fonctionnaire visé par une telle sanction, en ouvrant à celui-ci la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline lorsque l'autorité disciplinaire l'a informé de son intention de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Facultative et laissant une marge de négociation entre l'autorité disciplinaire et le fonctionnaire, cette procédure permettrait, en cas de contestation, de faire intervenir l'organisme paritaire comme médiateur. Elle pourrait présenter l'avantage de limiter le recours au juge administratif, la commission de recours étant présidée soit par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale, soit par un conseiller d'État dans les deux autres versants. Quel est l'avis de la commission ?

des sanctions de cette nature peuvent avoir des conséquences psychologiques particulièrement graves, y compris conduire à des actes irrémédiables. Nous en avons connu

On a coutume de prêter à la fonction publique beaucoup de défauts et les cas de passage de hauts fonctionnaires dans le secteur privé font la manchette des

implicite, faute d'instruction du dossier. Ce n'est évidemment pas acceptable. Le Sénat a formulé de nombreuses propositions depuis trois ans, par l'intermédiaire de la commission des lois ou de la commission d'enquête sur les mutations de la haute fonction publique

Nous allons vers un contrôle renforcé de la HATVP sur les cas les plus sensibles. Comme l'a dit Pierre-Yves Collombat en commission, l'enjeu n'est pas de contrôler un professeur qui ouvre une pizzeria ! Il

en confortant ses dispositifs d'investigation et en prévoyant une sanction pénale pour les agents qui ne seraient pas coopératifs. De même, elle refuse que le Gouvernement mette la main sur cette instance en tentant de reconstruire une commission de déontologie à l'intérieur même de la Haute Autorité. La HATVP est une autorité administrative indépendante et doit le rester. Ne tombons pas dans l'extrême inverse : la mobilité des agents vers le secteur privé n'est pas interdite,

Autant trop de postes faisaient l'objet d'un contrôle systématique à la sortie- c'est pourquoi nous restreignons ce champ en laissant au supérieur hiérarchique la possibilité de saisir en cas de doute la commission de déontologie

secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite, par cet amendement, apporter des précisions sur l'autorité à laquelle est transmise la déclaration d'intérêts et transposer le dispositif aux militaires. Dans le droit actuel, la déclaration d'intérêts est d'abord transmise à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui la communique ensuite à l'autorité hiérarchique chargée de procéder à l'analyse du contenu de la déclaration. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut parfois être directement le Président de la République ou le Premier ministre, ce qui ralentit évidemment le traitement de la déclaration. Aussi souhaitons-nous, afin de garantir une bonne gestion de ces déclarations d'intérêts, que le destinataire initial puisse être, selon le cas, soit l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit l'autorité hiérarchique de l'agent. Les modalités de transmission des déclarations entre ces deux autorités seront prévues par décret. Cette modification, je l'ai dit, serait également transposée aux militaires. L'amendement n° 244, présenté

Le projet de loi prévoit de rendre obligatoire pour les « fonctionnaires occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient

seuls « les fonctionnaires occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » seront contrôlés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en cas de création ou de reprise d'une entreprise. Cette disposition revient sur un apport important de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui avait étendu le contrôle de la Haute Autorité à tout fonctionnaire,

Une restriction du périmètre de contrôle à certains fonctionnaires est d'autant moins acceptable que c'est le Gouvernement qui déterminera par décret en Conseil d'État la liste des emplois assujettis à ce contrôle. Par ailleurs, à quoi servirait-il de créer une superstructure, fruit de la fusion de la HATVP et de la commission de déontologie de la fonction publique, si, plutôt que de lui octroyer les moyens nécessaires à ses missions,

Cependant, une telle saisine directe ne nous semble opportune que dans les cas où la saisine de la Haute Autorité est obligatoire. Dans les autres cas, la saisine doit demeurer une faculté relevant de l'appréciation de l'autorité hiérarchique, d'autant plus qu'elle ne peut intervenir que si l'avis du référent déontologue n'a pas permis de lever le doute sur la situation de l'agent. La saisine directe de l'agent ne paraît pas non plus adaptée dans le cadre du contrôle préalable à la nomination sur un emploi sensible, l'administration devant pouvoir maîtriser seule son processus de recrutement.

de la Haute Assemblée, notamment l'absorption de la commission de déontologie par la HATVP et l'institution d'un contrôle du rétropantouflage.

un cas, d'apprécier le dossier du fonctionnaire au moment de sa nomination ; dans l'autre, de prévenir les conflits d'intérêts au cours de l'exercice des fonctions. Le Gouvernement souhaite, dans certains cas, supprimer la transmission à l'autorité de nomination, ce qui constituerait un recul : celle-ci doit être suffisamment éclairée lorsqu'elle nomme un fonctionnaire à un poste sensible. En outre, le renvoi au décret semble inopérant : la liste des destinataires des déclarations d'intérêts constitue une garantie fondamentale pour les agents, et doit donc, de notre point de vue, être fixée dans la loi.

244, de Pierre-Yves Collombat, qui vise à établir la liste des corps soumis à déclaration d'intérêts. Cette liste serait, en réalité, moins large que celle qui serait qu'environ 7 500 agents publics sont aujourd'hui soumis à déclaration d'intérêts et que la liste fixée par décret inclut également des agents des collectivités territoriales, par exemple lorsqu'ils gèrent des marchés publics.

lui-même la HATVP. Il s'agit, notamment, d'éviter que l'administration ne bloque la mobilité de l'agent concerné en refusant de saisir le HATVP. Le Gouvernement fait un pas vers nous en acceptant cette disposition pour les emplois les plus sensibles, lorsque la saisine de la HATVP est obligatoire.

que celle que nous envisageons puisqu'elle ne concernerait que des hauts fonctionnaires. Or nous savons qu'un certain nombre de postes occupés par des agents de catégorie B ou C peuvent être tout aussi sensibles en termes de déontologie. C'est le cas des chefs de service chargés des marchés publics dans la fonction publique territoriale par exemple. Pour le reste, le Gouvernement ne partage pas

explication de vote. Comme vient de le dire ma collègue, nous ne sommes pas défavorables à la fusion du comité de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

pourraient être contrôlés. Or il n'y a pas que les hauts fonctionnaires qui peuvent être en situation de conflits d'intérêts. Il y en a d'autres, à tous les niveaux. Si la nouvelle autorité

un délai total de trois ou quatre ans pourrait en effet se révéler insuffisant. L'objectif est de permettre aux agents publics souhaitant se reconvertir professionnellement de le faire efficacement, dans l'intérêt général. Il n'est en effet pas satisfaisant ni pour les agents, ni pour les services où ils sont affectés, ni pour les administrés que des personnes effectuent leurs missions de service à contrecoeur, faute de passerelles acceptables.

Quel est l'avis de la commission ? Un fonctionnaire peut bénéficier d'un temps partiel pour créer son entreprise. Ce temps partiel est accordé pour une durée de deux ans, renouvelable pour un an, soit un total de trois ans. l'initiative de M. de Belenet, la commission a étendu ce délai à trois ans, en maintenant la possibilité de renouvellement pour une durée d'un an, soit un total de quatre ans. L'amendement de Mme Delattre, défendu par M. Labbé, vise à augmenter de nouveau ce délai, qui serait alors porté à quatre ans, renouvelable pour un an, soit un total de cinq ans. Il s'agit de laisser au fonctionnaire le temps de s'assurer de la viabilité de son entreprise, ce que nous pouvons tout à fait concevoir et soutenir. En outre, l'autorité hiérarchique pourra toujours refuser d'accorder ce temps partiel en raison des nécessités du service, ce qui paraît une mesure de bonne administration. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Pour les avis sur les projets de texte et les recommandations de portée générale concernant leur application, il est prévu de retirer du champ de compétence de la HATVP les premiers alinéas de l'article 25 du statut général qui détermine les obligations des fonctionnaires. En effet, la HATVP n'a vocation à se prononcer, comme la commission de déontologie avant elle, sur les principes déontologiques applicables aux fonctionnaires que dans le cadre de l'exercice de ses missions prévues aux articles 25 et 25 . Ces obligations vont au-delà de la seule question des conflits d'intérêts et n'entrent donc pas dans le champ de compétences de la HATVP : il s'agit des questions de dignité, de neutralité du service public, du principe de laïcité. La mention du dernier alinéa La mention du dernier alinéa de l'article 25 est conservée, afin de permettre à la HATVP d'examiner les chartes ou guides déontologiques soumis par les administrations, en particulier toute disposition en matière de prévention des conflits d'intérêts.

centraliser le contrôle effectif du respect des engagements de servir s'imposant aux anciens élèves des écoles supérieures du service public. Quel est l'avis de la commission ? Sur la question Sur la question éminemment importante de la pantoufle et de son remboursement, nous aurons un débat après l'article 16 , des amendements comparables ayant été déposés par le groupe socialiste et le groupe CRCE.

ira au-delà de la simple observation des documents qui pourraient lui être transmis. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement de Mme Taillé-Polian nous semble déjà satisfait par le texte. La commission a prévu, aux alinéas 67 à 71,

à haut niveau hiérarchique, communément appelés A+, constitue une difficulté pour l'établissement d'un système de contrôle déontologique satisfaisant du pantouflage.

leur exhaustivité étant toujours contestée. Un système alternatif pourrait être envisagé. Tel est précisément l'objet de cet amendement, qui vise à responsabiliser davantage l'autorité hiérarchique en lui confiant le soin d'apprécier

fin du contrat de travail conclu avec un employeur privé s'il est contraire aux dispositions que nous venons d'évoquer, impossibilité d'être recruté pendant trois ans pour un agent contractuel.

Pour plus d'efficacité, certains dossiers doivent remonter directement à la HATVP, pour éviter tout risque de collusion entre l'agent et son responsable hiérarchique. C'est notamment le cas pour les directeurs d'administration centrale et les directeurs généraux des services des grandes collectivités. à l'amendement n° 489 du Gouvernement. La commission a prévu une sanction pénale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'un agent public ne défère pas aux demandes de la HATVP. Il s'agit d'une sanction dissuasive, visant à assurer l'efficacité des contrôles de la HATVP et le suivi de ses réserves. Une peine similaire existe d'ailleurs pour les élus locaux. Dans l'affaire dite « Benalla », la commission d'enquête avait regretté que la commission de déontologie ne dispose pas d'outils de droit pénal pour renforcer ses contrôles. Quel est l'avis du Gouvernement ? Défavorable. La parole est à Mme

qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission- ces dispositions ne sont plus nécessaires, car la composition et les règles d'organisation de la HATVP relèvent de dispositions spécifiques.

Le Gouvernement est favorable à l'élargissement du périmètre des emplois, notamment dans les versants des fonctions publiques territoriale et hospitalière, pour lesquels les nominations sont soumises au contrôle systématique de la HATVP lors du retour ou de l'arrivée dans la fonction publique après une expérience dans le privé. Cependant, le champ de la rédaction adoptée en commission conduit à ce que tous les emplois supérieurs soient soumis au contrôle systématique de la HATVP, y compris certains emplois qui ne sont pas soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts. Ce champ trop large risque, selon nous, d'entraîner une dispersion du contrôle et d'empêcher que celui-ci soit suffisamment approfondi pour ce qui concerne les cas les plus sensibles. Or concentrer l'action de l'autorité indépendante sur les dossiers les plus sensibles constitue l'un des axes essentiels de la réforme proposée et adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale.

Le texte de l'Assemblée nationale était toutefois très timide : il concernait uniquement 228 emplois de la fonction publique d'État. La commission a substantiellement élargi ce périmètre. Elle a adopté un principe simple prévoir un contrôle du rétropantouflage pour tous les postes de direction que l'article 7 a ouvert aux agents contractuels. Avec l'amendement n° 485, le Gouvernement propose un compromis, et nous l'en remercions. Toutefois, notre rédaction nous semble plus efficace, car elle intègre, par exemple, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs des services déconcentrés et même les directeurs généraux des services des communes de plus de 40 000 habitants. Potentiellement, le champ peut paraître large, mais l'ensemble de ces postes ne sera pas occupé par des contractuels et l'efficacité des contrôles de la HATVP n'en sera pas affectée. En revanche, je suis ouvert sur le paragraphe I de l'amendement, qui permet au Gouvernement de fixer par décret en Conseil d'État le délai

en 2016, très peu a été fait pour endiguer l'influence des acteurs du numérique sur nos secteurs stratégiques et notre modèle démocratique. Pis encore, il semble régner au sein des hautes sphères de l'État une sorte de connivence à l'endroit des géants de l'internet. Les exemples ne manquent pas. Qui visez-vous ? En 2017, le directeur général de l'Arcep, le régulateur des télécommunications, a été recruté comme directeur des affaires publiques de Google, avant de remettre, deux ans plus tard, un rapport au Président de la République sur la régulation des plateformes, dans le cadre d'une mission effectuée auprès de Facebook. En avril 2018, c'était le directeur du numérique pour l'éducation au sein de l'éducation nationale qui s'apprêtait à rejoindre Amazon. Les géants du numérique ne se contentent pas d'aspirer les fonctionnaires des grands corps de l'État ; ils s'infiltrent dès les études supérieures pour attirer les étudiants des grandes écoles. Ainsi, en mars 2018,

à Sciences Po. Il y a urgence à établir un cordon sanitaire entre les grands corps de l'État et les entreprises privées. Il y va de notre souveraineté et de la protection de nos intérêts. Cet impératif passe par la formation et la sensibilisation des hauts fonctionnaires aux enjeux liés au numérique et par le renforcement du pouvoir et des compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Quel est l'avis de la commission ?

l'avis du Gouvernement ? Lors de l'examen des demandes des agents publics, la Haute Autorité doit étudier si l'activité envisagée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service public, si elle contrevient à tout autre principe déontologique et si elle ne risque pas de placer l'agent dans une situation de commettre un délit de prise illégale d'intérêts.

Selon les chiffres disponibles, 85 % des anciens élèves auraient « durablement » quitté l'État, mais pas définitivement, il faut le souligner. Toutefois, selon les corps d'origine, une part significative d'entre eux effectue des « passages

la mobilité vers le secteur privé est devenue, de façon coutumière, une étape de carrière, et ce avant même que la lutte contre les conflits d'intérêts ne devienne une préoccupation pour les pouvoirs publics, laquelle s'est notamment traduite à partir des années quatre-vingt-dix par l'adoption de la loi Sapin I. Pour autant, à présent que la lutte contre les conflits d'intérêts est devenue une priorité et qu'elle est nécessaire pour maintenir la confiance de nos concitoyens dans nos institutions démocratiques, il serait contreproductif de vouloir la concilier avec la préservation des intérêts personnels des anciens élèves de de l'ÉNA, en prévoyant dans le dispositif destiné à s'assurer que leur mobilité vers le secteur privé n'est pas préjudiciable à l'intérêt général que leur carrière doit être prise en compte.

bloquer la carrière d'un fonctionnaire, ce dernier étant alors contraint de partir à l'étranger pour se reconvertir, ce qui constitue une perte en capital humain non seulement pour l'administration, mais aussi pour le pays.

à mi-chemin entre le public et le privé. Aussi, le rapporteur a vraiment insisté sur un point d'importance : il faut créer une véritable direction des ressources humaines

d'un sujet d'actualité essentiel. Je forme le voeu que la mission menée par M. Thiriez et l'ensemble des contributions- rapport parlementaire, rapports des organisations spécialisées ou des organisations professionnelles et syndicales -nous permettront d'avancer dans les mois qui viennent.

Par conséquent, je suis assez surpris de la décision de la commission des lois d'avoir intégré cette disposition. Concernant un grand nombre de points,

Le délai applicable au nouveau contrôle préalable à la nomination dit « contrôle retour » sera, en revanche, déterminé par décret, comme le prévoit le paragraphe V de l'article 25 dans sa nouvelle rédaction. Ce délai sera inférieur à deux mois pour ne pas freiner le processus de recrutement des agents publics.

Cet amendement rejoint le texte adopté par l'Assemblée nationale, qui prévoyait que l'agent transmette une attestation annuelle à la Haute Autorité. Cette attestation semble toutefois particulièrement bureaucratique, et aucune sanction n'est prévue lorsque l'agent transmet une attestation erronée. erronée. La commission a préféré un autre système de contrôle, qui lui a semblé plus efficace : elle a renforcé les pouvoirs d'investigation de la Haute Autorité, qui organisera elle-même ses contrôles. Elle pourra ainsi hiérarchiser les cas les plus problématiques, disposera d'un pouvoir d'injonction et pourra, le cas échéant, saisir le juge pénal. La Haute Autorité devra rendre compte de ses contrôles dans son rapport annuel. Elle pourra également en publier directement les résultats. En conséquence, l'avis de la commission est défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? J'avais émis des l'avis du Gouvernement ? J'avais émis des réserves au sujet de l'adoption de ces dispositions par l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement se rallie aux propositions de la commission des lois du Sénat.

dernière peut donc parfaitement s'opposer au départ des agents, par exemple pour des raisons liées au bon fonctionnement du service public, et ce malgré un avis de compatibilité rendu par la Haute Autorité. Or le projet de loi prévoit désormais que tous les avis de la HATVP, y compris ses avis de compatibilité, s'imposent à l'administration.

Quel est l'avis de la commission ?

peut refuser le départ d'un agent pour le bon fonctionnement du service, même lorsque la Haute Autorité émet un avis de conformité sur cette mobilité. La commission y est donc favorable.

en cette matière précise, il nous paraît particulièrement nécessaire que soient soumis à la publicité les avis favorables assortis de réserves, sans quoi l'effectivité du contrôle de l'application de ces réserves serait considérablement affaiblie. Tel est l'objet de cet amendement

des avis de la HATVP. Je rappelle que la Haute Autorité n'aura à connaître que les cas touchant aux emplois les plus sensibles, du fait soit des fonctions occupées, soit du du niveau hiérarchique, les autres cas étant traités par l'autorité hiérarchique. Il faut également rappeler que ces sanctions concerneront des personnes se soustrayant délibérément

Du fait de leurs réseaux étendus et de leur fine connaissance de l'administration, il n'est pourtant pas rare de voir des hauts fonctionnaires retraités recrutés dans des cabinets d'affaires à des postes particulièrement lucratifs. Afin de permettre à l'administration de prononcer des sanctions plus dissuasives et proportionnées aux bénéfices tirés du non-respect des règles en vigueur en matière de prévention des conflits d'intérêts, nous proposons de supprimer le plafond de 20 % de retenue sur pension prévu à l'alinéa 63.

créent une entreprise, partent vers le secteur privé ou en reviennent. Il s'agit d'une clarification nécessaire : pour ces postes très sensibles, la saisine de la Haute Autorité doit être directe, sans marge d'appréciation de l'autorité Cet amendement s'inscrit dans le prolongement des conclusions d'une commission d'enquête sénatoriale désormais célèbre, la commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités